sur notre conception générale de la fiscalité et sur la place que doit y trouver l'impôt sur le revenu, qui est présumé le plus juste de nos impôts puisqu'il tient compte du revenu des assujettis. Nous avons souvent regretté qu'il n'occupe pas une place plus importante dans l'architecture de nos prélèvements obligatoires. En fait, c'est une véritable réhabilitation de l'impôt que nous entendons exprimer et une vraie progressivité que nous voulons mettre en oeuvre, afin de mieux faire vivre le principe selon lequel chacun doit contribuer en fonction de ses capacités. C'est la source même de notre concept républicain. Nous souhaitons donc rendre toute sa place à l'impôt sur le revenu et en accroître le rendement, et ce pour une raison simple : il est temps d'imprimer à notre droit fiscal une évolution majeure, en abandonnant les vieilles formules de taxation indirecte de la consommation qui pénalisent les ménages les plus modestes, et en rendant à l'impôt direct républicain toutes ses vertus. Le pari économique de ce gouvernement se trouve perverti par ce que l'on pouvait craindre, c'est-à-dire par le trop vif appétit des marchés financiers et boursiers en matière d'intérêts bancaires comme de dividendes. Mes chers collègues, en 1986, il y avait quatorze tranches d'impôt avec un taux maximal à 65 %. Aujourd'hui, nous en sommes à cinq tranches. J'aimerais que l'on nous réponde à la question suivante : la réduction

Tirant les enseignements d'une étude réalisée par l'IFOP pour le groupe Union Centriste, il tend tout d'abord à universaliser l'impôt sur le revenu en remplaçant le taux 0 % de la première tranche par un taux symbolique à 1 %. Peut-on, mes chers collègues, parler de « consentement à l'impôt » quand seulement 43 % des foyers fiscaux paient l'impôt sur le revenu ? Cette concentration de l'impôt sur les classes moyennes a d'ailleurs été doublement accentuée sous le quinquennat précédent, en 2014, quand François Hollande avait, par démagogie, supprimé la première tranche à 5,5 % et revalorisé par deux fois la décote. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise, dans un deuxième temps, à abaisser respectivement de 4 et de 2 points les deuxième et troisième taux du barème. Concrètement, nous proposons ainsi d'élargir l'assiette de l'impôt en soulageant du fardeau qu'elles supportent aujourd'hui les classes moyennes, à la fois trop riches pour bénéficier de nombreuses aides, mais trop pauvres pour faire appel à des conseillers fiscaux et optimiser leur facture fiscale. Cet abaissement significatif des taux serait d'ailleurs financé par la suppression de nombreuses niches fiscales, pour un surcroît de recettes fiscales de l'ordre de 6 milliards d'euros. Nous insistons sur ce point : il n'existe pas moins de 187 niches fiscales pour le seul impôt sur le revenu, soit un montant total de 33,3 milliards d'euros représentant quasiment la moitié des recettes nettes de cet impôt qui devrait, en 2019, peser 70,5 milliards d'euros. Coûteux budgétairement, ces dispositifs préférentiels constituent surtout une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, par une sorte de compartimentation et de « catégorialisation » des contribuables. Notez, mes chers collègues, qu'il est ici proposé d'abroger les seules niches dont l'effet incitatif ou social est jugé nul ou inefficient par l'Inspection générale des finances. Cette abrogation est plus que compensée par la baisse des taux et l'ajustement du barème. Ayons ce courage ! La question de la justice fiscale et de la lisibilité de notre système, on le voit ces temps-ci, est au coeur des soucis de nos concitoyens. Par cet amendement, il s'agit de répondre à la préoccupation d'un nombre croissant d'entre eux, en renouant avec l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, pour garantir notre pacte social et républicain, juge

L'impôt sur le revenu est, au fond, assez mal défini. L'un de ses défauts essentiels réside dans son assiette, par trop réduite, notamment au regard de la contribution sociale généralisée, qui s'apparente de plus en plus à un impôt sur le revenu de base. l'an dernier, du système du prélèvement forfaitaire libératoire, ou, a continué de miter cette assiette et le sens même de l'impôt, donnant une forme de traitement prioritaire aux revenus autres que ceux du travail. Cette étroitesse de l'assiette de l'impôt relativise toujours le débat que nous avons sur les taux d'imposition des tranches du barème. À nos yeux, la question du taux marginal est donc importante, sans être nécessairement déterminante. Il ne s'agit pas pour nous d'un dogme immuable de notre système fiscal, d'un signe fort qu'il conviendrait de préserver coûte que coûte : c'est tout simplement une nécessité. Nous nous attachons depuis de longues années à défendre et à illustrer le principe constitutionnel en vertu duquel chacun et chacune contribuent à la charge publique à proportion de leurs facultés. Je ne citerai pas ici les termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais les conditions sont peut-être réunies dans notre assemblée pour leur donner un relief particulier. Il est bon aussi que l'opinion publique puisse entendre les propositions que nous sommes en mesure de porter. La défense et l'illustration de ce principe passent, à notre sens, par un double mouvement de renforcement de la progressivité de l'impôt par le biais du barème et de rééquilibrage du traitement de la matière fiscale pour chacune des catégories de revenu. Comme je l'ai souligné hier dans la discussion générale, nous avons à réhabiliter les vertus de l'impôt. Cet amendement vise à favoriser le premier terme de ce mouvement en affirmant plus clairement la progressivité du barème, victime notamment de l'effet d'amortissement de la tranche centrale à 30 % qui traite pareillement des situations fort différentes. C'est aussi pour des raisons évidentes de rendement de l'impôt que nous avons déposé cet amendement. autant de recettes- nous voulons aider le Gouvernement à trouver de l'argent pour le budget de la Nation -qui permettraient de prendre en charge les dépenses utiles, de réduire les déficits et donc, dans les années à venir, de diminuer les impôts de tout le monde pour éviter à la France les travers de l'austérité.

de la tranche à 45 % du barème de l'impôt sur le revenu de 0,3 %, et non de 1,6 % comme c'est le cas pour les trois autres seuils. Pour des raisons d'économies budgétaires, le Gouvernement a décidé de sous-revaloriser, pour l'année 2019, les retraites, les allocations familiales et les aides au logement. logement. Sous l'hypothèse d'une inflation à 1,6 % en 2019, la revalorisation de ces prestations de seulement 0,3 % réduira le pouvoir d'achat de leurs bénéficiaires de 3,2 milliards d'euros. Le groupe socialiste et républicain s'oppose à cette sous-revalorisation, injuste socialement, et propose d'indexer ces prestations à hauteur de l'inflation. Pour financer en partie cette réindexation, en partie cette réindexation, nous souhaitons revaloriser de seulement 0,3 % le seuil de la tranche à 45 % du barème de l'impôt sur le revenu. Ce seuil passerait donc de 153 783 euros à 154 244 euros,

par nos concitoyens entre 2012 et 2016, on s'aperçoit que les deux derniers déciles des foyers fiscaux ont vu leur imposition

il est essentiel que chacun sache que les services qui sont apportés à la population ont un coût. Cela se mesure, notamment, par le consentement à l'impôt. En cela, nous relayons les préoccupations habituelles du groupe du RDSE et nous répondons

permettre aux classes moyennes de payer un peu moins d'impôt sur le revenu que ce qu'elles devraient acquitter normalement. Ils répondent ainsi à une partie des préoccupations des classes moyennes.

il n'y a pas que l'impôt sur le revenu qui finance les services publics. En effet, les personnes qui ne contribuent pas au titre de l'impôt sur le revenu payent beaucoup d'autres impôts : ...

pas trop de larmes de crocodile sur les couches moyennes et les hauts contributeurs à l'impôt sur le revenu : considérez plutôt certains renversements de situation ! Quand on parle des plus modestes, il faut savoir de quoi l'on parle.

de vote. Que M. le rapporteur général, qui s'est étonné de l'absence de l'amendement Caillaux relatif au rétablissement de la tranche à 5 % pour l'impôt sur le revenu,

Le groupe Union Centriste

de leurs moyens, doivent être mis à contribution. Le problème est que, en France, nous sommes les champions du monde des prélèvements obligatoires et que, en outre, ceux-ci sont

plus de 4 millions de foyers fiscaux bénéficient d'une demi-part de quotient familial amoindrie parce qu'ils sont constitués de personnes seules ayant élevé des enfants aujourd'hui majeurs, près de 200 000 personnes continuent de bénéficier du quotient dit « conjugal », car elles élèvent des enfants, et l'on compte plus de 9 millions de ménages ayant un ou des enfants soit gardés à domicile, soit en garde alternée, des ménages qui, la plupart du temps, sont d'ailleurs non imposables. Nous proposons donc de considérer et de traiter de la même manière l'ensemble des situations familiales, que les parents vivent seuls ou en couple.

sans parler de la mise sous plafond de ressources des allocations familiales. Avec ce gouvernement, la situation n'est guère meilleure. Voilà pourquoi les cosignataires de cet amendement proposent de porter le plafond du quotient familial de 1 551 à 1 750 euros

d'une importante notoriété. Ils inspirent admiration et reconnaissance à une majorité de Français. Ils représentent souvent une référence, voire un modèle, pour les jeunes générations.

imposer des personnes résidant à l'étranger sur la base d'un critère de nationalité est contraire aux règles de territorialité de l'impôt, qui sont fondées sur le critère de domiciliation fiscale en France, en application des articles 4 A et 4 du code général des impôts. Une imposition sur la base de la nationalité modifierait de manière substantielle les règles de territorialité en vigueur, prévoyant que les personnes non domiciliées en France n'y sont passibles de l'impôt que pour leurs seuls revenus de source française. Par ailleurs, en l'état actuel de la fiscalité internationale, une telle mesure serait rendue inopérante par les conventions fiscales qui nous lient à nos partenaires économiques. Le droit interne ne s'applique que sous réserve des conventions fiscales internationales, lesquelles ont force supérieure aux lois. Or, dans l'ensemble du réseau conventionnel, constitué d'environ 125 conventions fiscales qui couvrent la plupart de nos partenaires économiques, seul le critère de résidence permet à un État d'imposer les contribuables sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux. Il s'agit, ni plus ni moins, de la reprise des principes internationaux prônés par l'OCDE. Pour ces deux raisons, je demande le retrait de cet amendement.

En effet, il vise à rétablir le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficiaient les élus locaux avant la mise en oeuvre de la réforme du prélèvement à la source. Du fait de l'alignement sur le barème commun de l'impôt sur sont confrontés à d'importantes difficultés financières, alors que le mandat local reste plus que jamais le pilier de notre démocratie et de la confiance dans nos institutions.

habitants. La loi de finances pour 2017 a modifié le régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux en supprimant la retenue à la source libératoire. L'intégration

En outre, les indemnités des maires sont destinées à couvrir les frais qu'ils engagent dans le cadre de leurs fonctions. D'ailleurs, la quasi-totalité d'entre eux ne sollicitent pas le budget de leur commune pour se faire rembourser. Il s'agit d'une mesure de justice, la fonction d'élu local étant la plus prenante et la plus reconnue par nos concitoyens.

Guené. Les élus locaux, en particulier les maires des petites communes, assurent le lien de proximité dont les Français, spécialement dans les territoires les plus reculés, ont besoin. Ils sont disponibles à toute heure, et exercent leur et exercent leur tâche dans des conditions de plus en plus difficiles. Ils se sentent en effet délaissés par l'État et expriment aujourd'hui un profond découragement- beaucoup d'entre eux démissionnent.

nul au titre du prélèvement libératoire. Il faut savoir que ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire, mais sont la contrepartie de sujétions liées à leurs fonctions et à l'absence de remboursement d'une grande partie des frais qu'ils engagent. D'ailleurs, la circulaire du 15 avril 1992 précise

ou d'une fois et demie ce même montant en cas de cumul de mandats. Pour rappel, l'article 10 de la loi de finances pour 2017 a supprimé le dispositif de retenue à la source et a prévu l'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux au titre des traitements et salaires.

La fiscalisation des indemnités est-elle légitime ? L'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 658,01 euros par mois est-elle suffisante ? À ces deux questions, nous répondons par la négative, et nous refusons de céder à la démagogie anti-élus.

représentatif de frais d'emplois, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, d'une fois et demie ce même montant, soit 11 844 euros. Pour mémoire, le barème de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux était identique à celui du barème de l'impôt. L'abattement ne s'appliquait pas à défaut d'option pour la retenue à la source. la source. Ce système permettait aux élus locaux, en cas d'option pour le régime de la retenue à la source, de limiter la progressivité de l'impôt sur le revenu et de bénéficier de l'abattement. À titre d'exemple, les indemnités faisant l'objet de la retenue à la source et autres revenus des édiles soumis au régime applicable aux traitements et salaires pouvaient bénéficier, notamment, d'une double application de la tranche d'imposition à taux nul. Vous l'aurez compris, mes chers

conduirait à doubler, voire tripler, selon les seuils retenus, le montant de la déduction d'assiette dont bénéficient aujourd'hui les élus locaux. Madame Billon, les

ainsi que ce n'est pas demain que ce gouvernement, en dépit des belles proclamations et des incantations, s'attellera au grand chantier de la révision du statut des élus de France.

Excusez-moi de le dire de façon aussi forte, mais il est peut-être temps que ce gouvernement entende enfin les choses ! Hier, le Président de la République s'essayait à une séance de câlinothérapie avec les maires. Une sélection

L'idée n'est pas de protéger les uns ou les autres par un statut ; il s'agit de redonner sens à l'engagement public et à la cohésion nationale de tous les territoires.

proposons de réserver le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 1° de l'article 81 du code général des impôts aux seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu mensuel

Cela permettra d'avancer l'entrée en vigueur de ces dispositions, initialement prévue au 1 janvier 2020. L'article 58 sera en conséquence supprimé. L'exonération des aides des collectivités territoriales

et abordons avec esprit de responsabilité la situation de crise dans laquelle se trouve notre pays.

la contrepartie financière perçue par la personne âgée qui accueille à son domicile une personne- le plus souvent un étudiant -bénéficie déjà du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu prévu à l'article 35 du code général des impôts en faveur des personnes louant une partie de leur résidence principale pour un loyer raisonnable. La commission des finances et plusieurs sénateurs proposent de rétablir ce dispositif d'exonération, qui a été supprimé par l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse du Gouvernement. Il ne nous semble pas justifié de prévoir un dispositif d'exonération au seul bénéfice des personnes âgées. D'autres publics, telles

du bénéfice de la majoration de quotient familial, au seul motif qu'elle ne vivrait pas seules. Si votre amendement est adopté, madame Lavarde, il ne produirait aucun effet, l'article L. 631-17-1 du code de la construction

à tous les modes de recrutement, y compris dans le cadre d'une mobilité intragroupe. Ce régime s'applique à raison des rémunérations dues à compter du 1 janvier 2020 aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 16 novembre 2018. Il est proposé d'en étendre le bénéfice, pour les personnes dont la prise de fonctions

Les contribuables résidents fiscaux en Nouvelle-Calédonie qui reviendront en métropole à partir de 2019 ne bénéficieront pas de l'année blanche fiscale. Ils seront donc imposables aussi bien sur les revenus perçus en 2018 en Nouvelle-Calédonie que sur ceux qu'ils percevront en 2019 en métropole.

le bénéfice d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement dont le montant serait égal au montant de l'impôt sur le revenu néo-calédonien et plafonné à hauteur de l'impôt sur le revenu acquitté en métropole. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette proposition. En effet, dès lors que le prélèvement à la source sera mis en oeuvre, cela mettra fin à l'année noire que vivent actuellement les non-résidents l'année de leur départ de France. Grâce à la réforme, les contribuables qui s'expatrient n'auront plus à s'acquitter, dans le cours de l'année de leur expatriation, à la fois de l'impôt sur le revenu français au titre de l'année précédente et de l'impôt étranger, généralement prélevé à la source des revenus de l'année en cours. La situation des Néo-Calédoniens qui s'installeront en métropole après 2019 est identique à celle qu'ils rencontrent déjà aujourd'hui s'ils s'installent dans un autre pays ayant mis en place une retenue à la source. Il n'existe aucune justification à un tel avantage, qui remettrait en cause la logique même du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement mis en place dans le cadre du prélèvement à la source. En effet, les contribuables résidant en Nouvelle-Calédonie en 2018 n'ont pas supporté- et ne supporteront pas - de double contribution aux charges publiques au titre de l'impôt sur le revenu français l'année de leur retour en métropole. Ils sont placés dans une situation différente de celle des résidents de métropole et des départements d'outre-mer, dès lors que leurs revenus de l'année précédente ne supportent pas l'impôt Lors de leur retour en métropole après le 1 janvier 2019, ils seront soumis au prélèvement à la source relatif à l'impôt sur le revenu français au titre de leurs revenus perçus en métropole pour l'année en cours et devront acquitter, le cas échéant, le revenu néo-calédonien sur les revenus perçus l'année précédente, lorsqu'ils étaient résidents de Nouvelle-Calédonie. Il n'y a donc pas de double contribution aux charges publiques au titre d'un même impôt, mais bien deux régimes d'imposition distincts dont les modalités de recouvrement sont différentes, puisqu'elles s'appliquent à des revenus perçus ou réalisés au titre d'années différentes et profitent à deux collectivités différentes.

secrétaire d'État. Il s'agit d'exonérer de droits d'enregistrement les actes de notoriété suppléant à l'état civil pour les Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants, à l'instar du régime déjà appliqué pour les actes de notoriété destinés à suppléer les actes de l'état civil disparus à la suite de sinistres ou de faits de guerre. Cet amendement a été déposé tardivement devant votre assemblée, car il reprend

La commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition et a introduit dans le projet de loi de programmation de la justice les exonérations des droits d'enregistrement prévues par l'amendement dont nous débattons.

de programmation ? Je rappelle à cet égard que, contrairement à ce qui est indiqué ici dans l'exposé des motifs, il n'existe aucun monopole des lois de finances en matière de dispositions fiscales. Nous ne pouvons donc qu'être défavorables à un amendement de coordination avec des dispositions de fond que nous avons rejetées le mois dernier.

le Sénat vient de voter une augmentation de 125 % de la déduction fiscale des élus, qui revient à les exonérer d'impôt jusqu'à 1 500 euros par mois sur leurs indemnités. Je m'y opposerai évidemment en seconde lecture à l'Assemblée

ainsi libellé : La parole est à M. Roger Karoutchi. Le présent amendement vise à mettre le régime d'imposition des plus-values immobilières en faveur des opérations de logements en cohérence avec les choix opérés par ailleurs pour les outils de soutien à l'augmentation d'offre de logements. finances pour 2018, le Gouvernement avait souhaité les recentrer et leur donner de la visibilité, pour le logement neuf, dans les zones dites « tendues » : A , A et B1. Face à une demande soutenue, il est nécessaire de créer les conditions d'un choc d'offre qui, outre des simplifications réglementaires et une lutte accrue contre les recours abusifs prévus dans le projet de loi ÉLAN, nécessite la libération de plus de foncier. L'élargissement de ce dispositif exceptionnel d'abattement à la zone B1, proposé par le présent amendement, permet de rétablir la cohérence entre les choix opérés s'agissant du soutien de la demande de logement et de la libération de l'offre de terrains nécessaire pour y répondre. Quel est l'avis de la commission ?

de prendre en compte les frais qu'ils sont amenés à engager au cours de leur mandat. Il est proposé par notre collègue Claude Kern de permettre aux conseillers municipaux non défrayés de déduire fiscalement les frais de déplacement effectués dans le cadre de leur mandat.

financières décomposées en quatre volets, dont l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, l'IMAD. N'étant ni un loyer, puisqu'il n'y a pas de contrat de bail, ni une sous-location, cette indemnité, contrairement aux trois autres, n'a pas fait l'objet de précisions réglementaires quant à son régime fiscal. industriels et commerciaux, les BIC. Aucun de ces cas de figure n'est adapté à l'accueil familial. Sous réserve que le montant prévu entre les parties contractantes soit fixé « dans des limites raisonnables », dont l'absence de contours pose problème depuis des années,

mille accueillants familiaux sont concernés, prenant en charge, à leur domicile, des personnes âgées ou en situation de handicap. Ils ne sont ni des artisans, ni des commerçants, ni des industriels, encore moins des hébergeurs de touristes en chambre d'hôtes. Ils sont indispensables, au quotidien, à la prise en charge de personnes en difficultés du fait de l'âge ou du handicap. Il est donc proposé de supprimer cet article, dans l'attente de trouver une formule cohérente pour les hébergeurs

Elle constitue tout de même une solution de rechange intéressante pour les personnes âgées ou les personnes handicapées qui ne peuvent être maintenues seules à domicile et qui ne souhaitent pas aller dans un établissement spécialisé.

et que la mesure en faveur des chambres d'hôtes favorise les locations de type Airbnb, au détriment de l'hôtellerie. Si le Sénat ne peut que partager le souhait d'une meilleure évaluation des dépenses fiscales et d'une meilleure équité dans le secteur de la location la suppression de l'article 35 ne semble pas constituer une réponse adéquate. Cette mesure semble utile dès lors qu'elle incite à la mise à disposition, pour des étudiants ou des travailleurs saisonniers, de chambres à un tarif très raisonnable. C'est également un outil favorisant la cohabitation

concret et réel. Le président Retailleau l'a dit : on ne peut tripler ainsi le régime d'imposition des élus locaux, qui sont au plus près de la démocratie locale. Je note également que, l'année dernière, nous n'avons pas assisté au même niveau de prise de conscience et d'acuité du ministre de l'action et des comptes publics lorsqu'il s'est agi de réévaluer

cette initiative comme complètement irresponsable dans le climat actuel, en France et ailleurs. Quand le populisme- un mot dont on abuse parfois aujourd'hui

fécond, de trouver un point d'équilibre pour revenir sur une action passée dont on n'avait pas mesuré totalement et parfaitement les conséquences. Je trouve que la façon dont tout cela est fait,

nous avons mené un débat particulièrement riche et serein sur un sujet qui nous préoccupe tous.

que de revenir sur une fiscalité très défavorable-M. Retailleau et les autres orateurs l'ont rappelé -, en particulier pour les élus des toutes petites communes. Il ne s'agissait pas d'un privilège nouveau. Je suis,

lors de l'examen de l'amendement concerné, y compris, d'ailleurs, pour ce qui touche à la protection sociale et à la transition entre l'exercice d'un mandat ou d'une fonction exécutive locale et la reprise d'une activité professionnelle comme salarié ou dans la fonction publique, même si l'on sait que, dans le second cas, les choses sont un peu plus aisées du fait des dispositifs de mise en disponibilité ou de détachement. Nous